La séance est reprise. L’ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (projet n° 639 [2023 2024], je vous rappelle que ce scrutin s’effectuera depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle ci fonctionne correctement en l’insérant dans votre terminal de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, les agriculteurs n’attendent – hélas ! – plus grand chose aujourd’hui. Il s’articulait pourtant autour de plusieurs enjeux cruciaux pour l’avenir de notre agriculture.

et pour faciliter le plus possible les transmissions et la pérennité des exploitations. Je pense enfin à l’urgence d’alléger les contraintes et autres surtranspositions qui pèsent toujours plus au quotidien sur le secteur agricole. Hélas ! force est de reconnaître qu’au milieu de ces priorités, de nombreuses mesures pourtant essentielles n’ont pas été portées, par manque de courage. Aussi les agriculteurs n’attendent ils plus rien aujourd’hui de ce texte qui a perdu toute ambition.

Madame la ministre, vous n’êtes pas responsable de la situation : vous avez fait le job, dans la continuité des travaux parlementaires qui ont débuté il y a presque un an. Parmi les notions qui me paraissaient essentielles figurent les principes d’intérêt général et d’intérêt fondamental de la Nation, qui permettent de rétablir l’équilibre dans la hiérarchie des normes, afin de cesser d’opposer agriculture et environnement et d’éviter que les dispositions environnementales ne soient utilisées uniquement à des fins de blocage de tout projet. Il est temps, en effet, de retrouver du pragmatisme dans notre pays. Comme la Charte de l’environnement primera toujours, il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur une prétendue volonté des vilains législateurs, des vilains sénateurs, de faire de la régression environnementale un but. Je me suis battu pour que prévale la notion d’intérêt général majeur, pour que l’on ait le courage de définir des notions essentielles qui portent trop souvent à confusion et qui ont toute leur place dans la loi, comme la souveraineté agricole, la sécurité alimentaire ou encore la sécurité sanitaire alimentaire. J’ai échoué.

madame la ministre : transformer des milliers de kilomètres de bords de rivière en haies, ce n’est pas acceptable. On nous a imposé de légiférer sur des sujets accessoires comme la haie, le chien et même la laine.

Ce projet de loi ne sera qu’une étape. De toute façon, le coup était déjà parti, alors soyons positifs ! J’aime à rêver, madame la ministre, qu’il s’agit d’un nouveau départ pour l’agriculture, d’un changement d’air pour une ambition de souveraineté et de protection de l’environnement. Oui, un nouveau départ, face à une volonté clairement décroissante, poussée par de pseudo attentes inventées de toutes pièces par ceux qui attaquent la France.

au mieux trop ambitieuses, au pire mensongères, pour l’agriculture, rien ne bougera jamais non plus dans les autres secteurs. Cette période que nous vivons, avec la loi du plus fort qu’on tente de nous imposer en France et en Europe, devrait pourtant nous réveiller

de famines en disettes, de jacqueries en révolutions. La France a connu plus de périodes troublées par ce manque que de périodes de stabilité alimentaire, Faut il rappeler que, dans les années 1870, après la défaite de Sedan et la Commune, les Parisiens ont été contraints de manger les éléphants du zoo de Vincennes ?

gagné », nous l’avions « gagné » pour toujours ! Nous n’aurions plus besoin d’avoir peur, plus besoin de nous poser des questions sur notre capacité à produire

comme une atteinte à l’environnement et en faisant des paysans des assassins de la nature. Après des siècles d’asservissement aux seigneurs par les corvées, la taille,

qui subissent normes, règles, surtranspositions. Tant de paradoxes, de mesures parfois contradictoires, d’injonctions leur font perdre la tête ! Ils ont l’impression que l’on marche sur la tête, tant le bon sens paysan est attaqué. Comment leur dire qu’ils ne peuvent plus avoir les moyens de produire, car on les leur interdit, et que, dans le même temps, on laisse entrer des produits importés de pays voisins utilisant, eux, ces moyens interdits ? Comment ne pas les blesser au plus profond d’eux mêmes quand on leur dit qu’ils sont productivistes et que l’agriculture française est industrielle ? Ils vivent tout autre chose sur leurs exploitations familiales, dont les modes de production sont aux antipodes de ceux des produits que nous laissons entrer par nos accords de libre échange : les exploitations françaises comptent en moyenne soixante vaches, quand la viande que nous laissons entrer du Canada est produite dans des de 30 000 bovins. Qui peut raisonnablement comprendre cela ?

Après avoir trop voulu concentrer les politiques publiques sur la montée en gamme, par dogmatisme, et comme un enfant gâté qui oublierait le passé et qui arriverait à se convaincre de ses propres forfaitures, nous allons enfin ériger la souveraineté alimentaire en intérêt fondamental de la Nation et veiller à ce qu’elle ne régresse plus. Oui, la souveraineté alimentaire est le seul moyen de nourrir son peuple sans avoir à recourir massivement aux importations – et en prenant bien soin de nourrir toutes les bouches, tant de ceux qui ont les moyens que de ceux, les plus pauvres, qui sont obligés d’arbitrer entre leurs achats.

commerciale française, vins et spiritueux compris, a encore chuté de 1,6 milliard d’euros cette année. Il ne restera bientôt plus rien de cet excédent. cet excédent. Ce fleuron de l’économie française exporte non seulement une simple denrée alimentaire, mais aussi une histoire de paysans, un savoir faire mondialement reconnu, un terroir et le labeur de tous ceux qui cultivent et élèvent avec une passion sans pareille. Ces mauvais résultats nous obligent. Nous ne pouvons plus regarder passivement décliner la France agricole, car c’est notre histoire que nous injurions ; c’est notre patrimoine que nous dilapidons ; c’est notre survie que nous condamnons en laissant notre agriculture s’amenuiser, avec le risque de la voir disparaître. Cet après midi, je veux avoir une pensée toute particulière pour les producteurs de noisettes, de kiwis, de cerises, de pommes, de poires, de bananes, d’endives, de betteraves, de pommes de terre, mais aussi pour les éleveurs de porcs et de volailles. Et la liste n’est pas exhaustive, tant le problème est grand ! Alors – c’est vrai pour reprendre la rhétorique de certains, changeons de modèle ! Oui, mais changeons de modèle de pensée ! Rappelez vous la phrase de Jean Jacques Rousseau : « L’agriculture est le premier métier de l’homme : c’est le plus honnête, le plus utile et, par conséquent, le plus noble qu’il puisse exercer.

ce projet de loi aura traversé toutes les saisons. Présenté au printemps dernier en Conseil des ministres, il a ensuite subi la sécheresse législative de l’été 2024, avant d’être laissé en jachère pendant un automne très instable. Ce parcours exceptionnellement long est sur le point de s’achever, à la fin d’un hiver particulièrement fertile pour les sujets agricoles dans notre hémicycle. Après six journées de débats passionnants, intenses,

Je pense ainsi à la mise en place du contrat territorial de consolidation ou de création de formation, qui permettra d’augmenter le nombre de jeunes formés par la voie initiale scolaire dans les établissements de l’enseignement agricole technique. J’ai également en tête l’article 5 du projet de loi, qui prévoit la création du bachelor agro, un diplôme qui sera reconnu au niveau bac+3. De plus, la mise en place du réseau France installations transmissions, ou France Services agriculture, est prometteuse et sera – j’en suis sûr un des éléments essentiels de ce texte, que les agriculteurs apprécieront au moment d’acquérir ou de céder leur exploitation. Grâce à ce nouveau guichet départemental unique, l’État doit offrir un nouveau service public accessible de qualité avec l’appui des chambres d’agriculture. pas le dispositif d’aide au passage de relais créé au Sénat : une aide transitoire de 1 100 euros par mois pendant une durée maximale de cinq ans avec prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite de l’exploitant et des membres de sa famille qui participent aux travaux. Pour renouveler les générations, nous devons également donner un coup de pouce financier aux retraités de demain. Avec cet engagement, ce nouveau réseau, le bachelor agro et le contrat territorial, nous semons des graines qui germeront rapidement dans l’intérêt du renouvellement des générations.

Des premiers accords de libre échange aux négociations avec le Mercosur, en passant par la pandémie de covid 19, nous avons toutes et tous constaté l’importance de la notion de souveraineté, qui plus est lorsqu’il s’agit de nourrir la France. Mais force est de le constater, face aux enjeux de transition liés à l’environnement, à l’environnement, le monde agricole a parfois le sentiment d’être relégué au second plan, alors que, dans le même temps, nous voulons que l’agriculture soit une fierté française. Il est donc nécessaire d’encadrer juridiquement le sujet, non pas pour placer l’agriculture au dessus de l’environnement, mais pour mieux équilibrer la balance. Nous atteignons, je pense, une forme d’équilibre, puisque nos débats ont penché en faveur d’une souveraineté alimentaire érigée au rang d’intérêt fondamental de la Nation, avec un principe de non régression. Enfin, nous voterons ce projet de loi, parce que nos débats en séance ont permis d’introduire des mesures essentielles. Je veux bien évidemment aborder l’évolution du cadre juridique applicable à la haie. Nous avons, je crois, retenu une définition équilibrée. J’ajoute que l’adoption de mon amendement permettra d’exclure de ce qui relève d’une destruction de haies la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation « chemin rural ». En l’absence d’une telle précision, la rédaction de l’article 14 risque de constituer un obstacle majeur à la réouverture des chemins ruraux, en imposant, d’une part, le respect d’une procédure qui, à la base, n’est pas prévue pour ce cas et, d’autre part, la compensation du linéaire détruit par les communes, ce qui sera très difficile.

Telles sont les principales raisons qui poussent notre groupe à se prononcer en faveur de l’adoption de ce projet de loi. Nous savons d’avance que ce texte seul ne réglera pas l’ensemble des problèmes rencontrés par nos agriculteurs. il permettra de poser des fondations solides au sursaut patriote agricole que je souhaite pour notre pays et sera complété, je l’espère, par d’autres textes pour en combler les angles morts. Je fais ici référence au revenu des agriculteurs ou au sujet du foncier. Mes chers collègues, vous le savez, dans quatre jours, le Salon international de l’agriculture sera lancé. Si l’adoption définitive du texte avant ce lancement reste incertaine, ce qui, en revanche, est sûr et certain, c’est que j’agirai autant que possible pour que la commission mixte paritaire puisse être conclusive. dès cet après midi l’occasion de retisser ensemble le lien de confiance avec celles et ceux qui font de l’agriculture une fierté française et faisons en sorte que ce texte soit adopté le plus rapidement possible. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après de multiples retards, la grande loi agricole promise au mois d’avril 2022 par Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle, est enfin sur le point de voir le jour. l’adjectif « grande » est de trop : entre les intentions de départ et le texte présenté aujourd’hui, le contexte et son contenu ont radicalement changé. Pourtant, nous partons du même constat : le déclin de la puissance agricole française. L’enjeu derrière cela, c’est la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire et du revenu des agriculteurs. Si l’intention initiale – moderniser notre modèle de production pour regagner en compétitivité – demeure, la nette atténuation de l’ambition écologique invite à la plus grande vigilance. à coup de « pragmatisme » et d’ambition en matière de compétitivité, le texte qui nous est présenté aujourd’hui s’est éloigné d’un de ses objectifs initiaux : rebâtir la souveraineté alimentaire de la France en répondant notamment au défi du changement climatique. L’agriculture est pourtant l’un des secteurs d’activité les plus sensibles à l’évolution du climat et les plus dépendants du fonctionnement des écosystèmes. L’objectif d’une agriculture économiquement et écologiquement viable, rémunératrice, diversifiée, durable et répartie sur l’ensemble du territoire doit prédominer et servir de mise en garde contre la stérilité de l’opposition entre agriculture et environnement. Or je n’ai pu que constater et déplorer au cours des débats la crispation de certains lorsqu’il était question de transition vers une agroécologie et d’adaptation au changement climatique. Au delà de ces constats, plusieurs interrogations me viennent à l’esprit. J’espère qu’elles trouveront une réponse équilibrée dans la commission mixte paritaire. D’abord, le diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles, désormais beaucoup plus économique qu’environnementale, avec ses six modules mobilisables indépendamment les uns des autres, n’est plus obligatoire. Certes, ces derniers seraient gratuits en cas de mobilisation lors de périodes clés d’un projet agricole, c’est à dire en début ou en fin de parcours. Néanmoins, leur réalisation sur la base du volontariat, mettant par conséquent fin à l’obligation de leur réalisation, me pose question. La logique incitative visée par le texte peut ne pas être suffisante ; elle nous plonge dans une certaine opacité. Seul un engagement contraint permettrait de répondre aux conditions d’installation viables dans le temps, notamment du point de vue de la performance agronomique des sols de l’exploitation. le rappelle, en soixante ans, nos sols ont perdu 80 % de leur matière organique et entre 70 % et 90 % de leur population bactérienne et fongique. Leur tassement s’est irrémédiablement accentué. Installer des jeunes sur des sols qui ne fonctionnent pas dans un système figé et de plus en plus intégré dans la chaîne de distribution est une erreur. Et le faire en connaissance de cause est, à mon avis, irresponsable. Je regrette le rejet en séance publique de l’attribution d’une septième mission à l’enseignement agricole. Il était envisagé d’intégrer au programme de la formation initiale et continue agricole des modules sur les tâches administratives auxquelles les agriculteurs feront face dans leur carrière. le rappelle, 20 % à 25 % du temps de travail d’un agriculteur est consacré à des tâches administratives. Certains lycées agricoles de mon département ont relevé un tel manque. Cet enjeu doit être désormais une nécessité de la formation agricole. Or l’État ne joue pas encore pleinement son rôle et se doit de mettre en œuvre une vraie politique publique en matière d’accompagnement et de sensibilisation aux réalités du métier d’agriculteur. ci sont encore trop floues pour les principaux concernés, et elles le sont encore plus aux yeux de nos concitoyens. Faire de notre agriculture une grande cause nationale n’est pas une incantation. Ou bien estimez vous que la santé mentale des jeunes aussi relève du superfétatoire Recréer un lien entre l’urbain et le rural, le citoyen et l’agriculteur, le travailleur de la terre et le jardinier du dimanche, pour sensibiliser chacun sur les atouts de notre agriculture, au delà de nous nourrir et de maintenir nos paysages, est une nécessité, ne serait ce que pour susciter de nouvelles vocations. À ce titre, si ce texte cherche à apporter plusieurs réponses au défi du renouvellement des générations, que ce soit en fixant des objectifs ambitieux en matière de hausse du nombre d’élèves de l’enseignement agricole, notamment par une meilleure visibilité et attractivité de ses filières, ou en renforçant la pertinence de la lisibilité du parcours d’installation et de transmission des exploitations agricoles par la mise en place d’un guichet unique, une absence se fait remarquer : celle de l’accès au foncier agricole. Aucune disposition concrète ne permet de libérer du foncier agricole utile, afin de faciliter la politique d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations. Madame la ministre, vous vous êtes engagée pendant le débat sur un projet de loi. Mais ne pensez vous pas qu’un travail en amont serait nécessaire ? Je pense par exemple à une mission sur le foncier agricole. Pourtant, ce projet de loi s’attache à dessiner un cap clair pour l’agriculture française, fondé sur une triple ambition consacrer le principe de souveraineté alimentaire, créer des conditions d’installation viables dans le temps et passer de réflexes de suradministration et de sanctions à une dynamique d’information et d’incitations. La dépénalisation de certaines atteintes environnementales en l’absence de négligence grave ou d’intentionnalité m’interroge aussi, même si je reconnais une volonté de simplification.

L’équilibre consistant à faire coïncider les objectifs de souveraineté, de simplification normative et de compétitivité où l’enjeu climatique et la préservation de la biodiversité seraient centraux ne me semble pas respecté dans ce texte, et ce malgré vos efforts, dont je vous remercie,

en plus d’avoir été de nouveau amputée de 200 millions d’euros en commission mixte paritaire, nous a déjà prouvé que la planification écologique était la variable d’ajustement. C’est désormais à la commission mixte paritaire – vous l’avez compris, nous y tenons beaucoup – de trouver un équilibre satisfaisant pour avancer vers un modèle d’agriculture protecteur de l’environnement et plus résilient en attendant d’être plus rémunérateur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous votons aujourd’hui un projet de loi important, aboutissement de plusieurs mois de discussions pour l’avenir de notre agriculture. Ce texte s’inscrit dans un contexte où les attentes des agriculteurs sont plus que pressantes, à quelques jours du salon de l’agriculture, qui débutera à la fin de cette semaine. Il est essentiel de se rappeler que, derrière chaque chiffre et chaque mesure dont nous avons débattu dans cet hémicycle, il y a des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à nourrir notre pays. Ces travailleurs de la terre sont autant d’individualités avec leurs aspirations, leurs frustrations et leurs espoirs. Un des slogans les plus entendus en 2024 a, à lui seul, illustré le profond malaise des agriculteurs : « On marche sur la tête. » Ce cri de désespoir, accompagné d’une opération de retournement de panneaux de communes, a perduré cet hiver sur fond de négociations commerciales avec le Mercosur. Ce slogan suffit à résumer et à dénoncer les injonctions contradictoires adressées à l’agriculture. Les agriculteurs expriment ainsi une quête unanime de reconnaissance, qui se traduit sur le terrain des politiques publiques

Comment demander à nos agriculteurs de produire de manière exemplaire tout en laissant d’autres producteurs étrangers les concurrencer dans des conditions moins contraignantes ? Nous donnons les moyens à d’autres de produire, mais non pas à nos propres agriculteurs, et ce sans garantir une homogénéisation des normes de production à l’intérieur du marché unique ou au sein des accords commerciaux. Les agriculteurs souffrent ainsi d’une suradministration toujours plus importante et passent en moyenne neuf heures par semaine à effectuer des tâches administratives. Par ailleurs, ils aspirent à une concurrence « à armes égales ». Face à un marché mondial ouvert, ils demandent une harmonisation des normes entre les États européens et une « exception agricole européenne vis à vis des pays tiers qui ne respectent pas nos standards afin de rester compétitifs. À leur niveau, les réglementations françaises aggravent parfois ces inégalités de concurrence. Ainsi, 37 % des agriculteurs évoquent un « abandon » et un « système à bout ». Cela témoigne du désespoir face à un échelon national qui semble se retourner contre eux au lieu de les soutenir. Ce texte ne doit rien au hasard. Il s’inscrit dans un contexte particulier : celui d’une agriculture en difficulté, dont les maux ont été identifiés bien en un amont par les nombreux travaux menés par le Sénat ces dernières années. En effet, dès 2022, la commission des affaires économiques alertait le décrochage de la ferme France. Cette situation, pourtant déjà préoccupante, s’est alors aggravée. En témoigne la diminution de l’excédent commercial agroalimentaire de la France, qui est passé de 12 milliards d’euros à 4,9 milliards d’euros entre 2011 et 2024. Ce qui manque particulièrement dans ce texte, c’est un véritable volet économique adapté aux enjeux de compétitivité du secteur. Bien que l’aspect environnemental soit primordial, il ne faut pas oublier que le développement durable de l’agriculture repose sur un triptyque équilibré entre l’humain, l’économique et l’environnement. C’est là la différence des visions qui se sont confrontées dans cet hémicycle. Or, aujourd’hui, ce texte semble accorder une place prépondérante au pilier environnemental en négligeant les autres aspects. Si l’agriculture durable doit intégrer des normes écologiques, elle doit également offrir aux agriculteurs les moyens de vivre dignement de leur métier, avec des revenus stables et des perspectives économiques claires pour les générations futures. Néanmoins, ce projet de loi, mes chers collègues, n’est pas sans avancées. Il contient plusieurs éléments qui vont dans la bonne direction pour soutenir les agriculteurs. Je retiens notamment une philosophie d’expérimentation intéressante, avec, par exemple, l’article 10 , qui instaure un droit à l’essai et permet aux agriculteurs d’expérimenter de nouvelles pratiques sans crainte des sanctions en cas d’échec. Je pense également à l’article 13 , qui introduit un droit à l’erreur permettant de prendre en compte les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de nouvelles normes sans pénaliser les agriculteurs de bonne foi cherchant simplement à s’y conformer. Faisons confiance à nos agriculteurs et laissons les innover dans leurs pratiques ! Par ailleurs, ce texte contient également des mesures de bon sens, ce bon sens auquel nous n’avions de cesse de nous référer pendant nos débats. Je pense par exemple à l’article 10 A, Vivea et le compte personnel de formation (CPF), permettant aux agriculteurs d’accéder plus facilement à des formations adaptées à leurs besoins, notamment dans leurs projets d’installation. Je pense également à l’article 3 , favorisant les collaborations entre centres d’apprentissage et centres de formation continue, ou à l’article 11, qui soutient la création de groupements d’employeurs. Ces mesures pragmatiques permettent d’alléger les charges administratives des exploitations et d’en améliorer la gestion des ressources humaines. Enfin, les articles 1, 2 et 8 encouragent l’installation des femmes dans l’agriculture. Loin d’être anecdotiques, ce sont de réelles avancées pour féminiser notre agriculture quand on sait que les agricultrices sont 100 000 aujourd’hui contre un million à la fin des années 1960. Pour autant, à la suite de l’examen sénatorial du projet on constate un effet de rattrapage. En effet, ce texte gouvernemental est utilisé comme véhicule législatif balai pour y intégrer diverses qu’il s’agisse d’eau et d’assainissement, de gestion de haies, de santé des sols, etc. Ce n’est pas une pratique nouvelle, mais cela reflète le fait que, dans un contexte politique incertain, un gouvernement légifère par propositions de loi et que des parlementaires cherchent à tordre le bras de l’article 45

Cependant, certains points de ce texte nécessitent des ajustements. D’une part, ce projet de loi est censé donner une impulsion pour l’installation et la transmission des exploitations agricoles pour les dix prochaines années. Or l’on voit déjà poindre des débats complémentaires sur le foncier et les revenus agricoles. Ces débats sont pourtant au fondement de l’équilibre des agriculteurs et de leurs exploitations. D’autre part, l’examen s’est parfois concentré sur des points sémantiques ou très ou très indirectement liés à la souveraineté alimentaire, qu’il s’agisse de l’article 10, relatif au nom du futur guichet unique, ou de l’article 14, à propos du cadre législatif portant sur les haies. Cela Cela interroge à la fois sur les irritants parfois absurdes, mais également sur l’inflation normative. Mes chers collègues, malgré des points d’amélioration, ce projet de loi représente un pas en avant pour l’agriculture française. Il permet de lever des obstacles bien identifiés et d’offrir de nouvelles marges de manœuvre aux agriculteurs, afin que ces derniers puissent rivaliser sur un pied d’égalité avec leurs voisins européens et mondiaux. La version sénatoriale de cette loi repose sur de nombreux travaux législatifs de notre chambre

les hasards du calendrier ont voulu que nos débats au Sénat se rapportant à l’agriculture coïncident avec les élections aux chambres d’agriculture. Dans le strict respect d’un scrutin qui appartient en propre aux agriculteurs et aux salariés agricoles eux mêmes, et sans faire dire au scrutin autre chose que ce qu’il signifie, on peut noter que la colère continue à s’exprimer dans le monde paysan. Et c’est normal, car, en l’occurrence, le revenu n’est jamais garanti d’avance, en raison de l’incertitude permanente qui plane sur l’avenir des filières et sur la fixation des prix agricoles.

La loi d’orientation agricole aurait pu constituer la bonne occasion pour fixer un certain nombre d’objectifs, infléchir un certain nombre d’orientations et se donner ainsi les moyens d’œuvrer dans le sens du développement durable de notre agriculture. Il n’en est rien ; bien au contraire ! Les principales dispositions retenues dans ce texte consistent à considérer que la planche de salut de notre agriculture résiderait dans une recherche de compétitivité à tout prix, permettant une intensification de la productivité en s’affranchissant d’un certain nombre de contraintes réglementaires et même de préconisations scientifiques. Cela a pour effet d’alimenter une dualité entre la société et les agriculteurs. Certes, les excès de paperasserie et les lourdeurs administratives exaspèrent les agriculteurs, et l’on peut comprendre leur agacement. Il convient donc de lever de telles lourdeurs. Mais cela ne doit en aucun cas servir de prétexte pour en rabattre sur un certain nombre de prescriptions. Sachons toujours nous rappeler

Nous avons également relevé que, pour répondre à ces objectifs d’intensification des productivités, les options retenues tendent à mettre à mal les potentialités que recèdent l’agroécologie, l’agriculture biologique et l’enseignement de ces disciplines. Pipeau ! En outre, ces orientations créent un clivage tendant à opposer agriculture et écologie. Certes, l’agriculture de production est une activité humaine indispensable à la survie de l’humanité. Mais, pour continuer à assurer cette mission, il est indispensable de se remettre en question. Le modèle de développement à promouvoir ne peut, par exemple, pas être celui de l’industrialisation de l’engraissement des bovins, comme on le pratique par exemple au Texas, avec des unités de 75 000 têtes auxquelles on fait gagner

: « La terre est faite pour être entre les pattes des animaux ! » Nous sommes en effet dans des régions d’élevage. Si la société a perdu un peu confiance dans l’industrie agroalimentaire, nos concitoyens croient encore à la sincérité des éleveurs, qui travaillent au contact de la nature. C’est là aussi un élément de motivation pour façonner nos paysages, nos haies, nos talus, nos bocages.

La crise agricole est structurelle, elle révèle les limites d’un modèle insoutenable. C’est votre bilan ! Ce projet de loi aurait dû être le texte d’une refonte de notre modèle vers la transition agroécologique, une transition indispensable pour assurer un accompagnement des agriculteurs face aux défis immenses qu’entraînent le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la chute sans fin du nombre d’agriculteurs. Mais ce texte s’emploie à détourner la colère des agriculteurs des véritables responsables.

Il ne relève ni le défi de l’accès au foncier et de l’accaparement des terres ni celui, pourtant majeur, de l’élevage, qui est fragilisé. Il renvoie ces sujets fondamentaux à de futures lois. lois. Il ne répond pas non plus à l’aggravation des inégalités entre les mondes agricoles, où il n’y a pas grand chose de commun entre les grands céréaliers exportateurs, qui captent la majorité des aides publiques de la PAC, et les petites exploitations en polyculture, élevage ou maraîchage, qui nourrissent nos territoires, entretiennent les paysages et se partagent ce qu’il reste des aides. En refusant de donner un cap vers la transition, en refusant le pluralisme, vous renforcez en vérité l’évolution vers l’agro industrie et vous nous menez à une impasse. En effectuant une lecture fallacieuse des données agricoles, en niant les faits scientifiques, vous prenez une lourde responsabilité. Concernant l’examen du texte en séance publique, nous déplorons l’absence manifeste de volonté de compromis pendant ces six jours de débats. Aucun apport réellement structurant venant de la gauche n’a été adopté. C’est assez rare que les propositions des groupes d’opposition soient aussi peu considérées et nous le regrettons. Quasiment tous nos amendements ont été rejetés, qu’il s’agisse de mieux réguler le foncier – sujet mis à la trappe par le couperet arbitraire de l’article 45 de la Constitution –, de mieux former les agriculteurs de demain, notamment sur les enjeux de transition agroécologique,

Une seule éclaircie : l’intégration de la proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie, adoptée à l’unanimité. Concernant l’article Concernant l’article 1, votre définition de la souveraineté alimentaire ne se fait que sous le prisme de la compétitivité. Une souveraineté biaisée qui, en renforçant une volonté exportatrice, ne respecte pas la souveraineté des autres pays.

Toutes les références et tous les objectifs relatifs à l’agroécologie et à la bio ont été supprimés, tant dans les orientations des politiques publiques que dans les objectifs de la formation et de l’enseignement professionnel agricoles. Ce texte ignore donc les grands défis du XXI siècle. L’agriculture doit faire sa mue pour s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Elle émet 19 % des gaz à effet de serre et doit prendre sa part dans les impératifs de réduction. Rien dans ce texte ne traduit cette ambition.

est une attaque délibérée contre la biodiversité et la santé humaine. Ce dispositif ne devrait d’ailleurs pas tenir devant le Conseil constitutionnel. l’enseignement, enjeu central pour assurer le renouvellement, le cap n’est pas le bon et les moyens ne sont pas au rendez vous. Le bachelor agro que vous souhaitez axer sur les compétences managériales et entrepreneuriales pour formater de futurs agriculteurs à une vision concurrentielle et productiviste est un entonnoir vers l’endettement et l’agrandissement. La création et la reprise d’activités agricoles sont pourtant de formidables opportunités pour engager la transition du secteur, mais le texte ne fait l’objet d’aucune mesure concrète pour soutenir des installations, d’abord agroécologiques, car en cohérence avec les attentes d’une majorité de futurs agriculteurs. La priorité aurait dû être d’établir un véritable pluralisme au sein du futur réseau France installations transmissions et dans la composition des instances associées à sa gouvernance. Mais vous êtes restés sourds à cette nécessité. Il en est de même pour le diagnostic modulaire, un outil initialement consacré à la transition : vous l’avez dévoyé, puisqu’il est désormais centré sur le modèle économique des exploitations, mettant de côté les aspects sociaux et environnementaux. Sur l’article 13, nous sommes toujours sidérés par ce qui constitue l’une des pires régressions en matière de droit de l’environnement de ces dernières années. En allant vers une véritable dépénalisation de la destruction d’espèces protégées choisie ne concerne pas seulement le secteur agricole ! –, le texte issu du Sénat est contraire à la directive européenne sur la protection de l’environnement. Les plus hautes instances juridiques censureront vraisemblablement ce dispositif. Comptez sur notre vigilance et notre mobilisation ! À l’article 15, c’est la concertation et le débat qui sont amputés pour mieux industrialiser le monde agricole. Avec ce texte, nous sommes à contresens de l’Histoire et de l’urgence écologique, mais en phase avec le plan social en cours. C’est pourquoi le groupe Écologiste Solidarité et Territoires votera résolument contre. Non, les décisions politiques ne peuvent pas être influencées par les voix les plus bruyantes ou les intérêts d’une minorité au mépris du pluralisme et de la démocratie. Face aux réalités climatiques, sanitaires et environnementales, nous continuerons de défendre l’intérêt général et des réponses structurelles pour la rémunération des paysans et la préservation de notre capacité à produire demain sur des sols vivants. Bravo La parole est à M. Jean Claude Tissot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

nous voilà au bout, ou presque, du parcours législatif tumultueux du projet de loi d’orientation agricole. Après de longs mois d’attente, six jours de séance, trente cinq heures de débats et environ huit cents amendements examinés, quel est le résultat ? Nous avions reçu de l’Assemblée nationale un projet bavard et imparfait, n’apportant guère de réponses concrètes au malaise agricole. Si, madame la ministre ! Comme nous pouvions le prévoir, et dans une connivence permanente avec le Gouvernement, les rapporteurs ont donné une connotation encore plus économique et libérale au projet de loi. Nous allons donc sortir du Sénat avec une loi fleuve, floue, dangereuse pour l’environnement et qui met en avant une certaine idée de l’agriculture, dépassée depuis longtemps. D’ailleurs, ne devrait on pas parler plutôt de « loi d’orientation pour une agriculture productiviste » ou encore de « loi d’orientation pour une agriculture passéiste » Vous avez, messieurs les rapporteurs, madame la ministre, modelé un texte parfaitement comme vous le souhaitiez à coups de dogmes pro industrie agroalimentaire et anti environnement. Monsieur le rapporteur Laurent Duplomb, vous avez indiqué que ce texte ne serait pas le Grand Soir de l’agriculture. Nous voilà d’accord À travers ce texte, vous perpétuez la trajectoire agro industrielle de l’agriculture, tournée vers le gigantisme, l’accaparement des terres, le productivisme à tout va. Nous soutenons deux modèles qui s’opposent frontalement et je ne vois même pas où nos positions pourraient se rapprocher Finalement, au terme de débats à sens unique, ni la crise sanitaire, ni la crise environnementale, ni la crise économique, ni – surtout ! – la crise du renouvellement des générations ne se voient proposer de réponses à la hauteur. Et au bout du compte, ce seront les paysans qui paieront la note – comme toujours Après le moment agricole que nous avons traversé et à quelques jours de l’ouverture du salon de l’agriculture, je le confesse, je suis très inquiet. Je suis inquiet pour l’avenir de notre agriculture de manière générale. Qui peut croire que le modèle hyperproductiviste, avec la crise perpétuelle dont il est la source, est attractif pour de jeunes actifs agricoles ? Le modèle consacre un entre soi d’exploitations gigantesques et intransmissibles. On peut nous accuser de grossir le trait, mais regardez où nous en sommes aujourd’hui.

qu’un pansement sur une jambe de bois. Il ne sera pleinement utile que lorsque nous nous engagerons sur la voie d’exploitations à taille humaine. Je suis aussi inquiet pour les agriculteurs et pour leur santé. Dans la continuité des débats tenus ici ces dernières semaines, le texte revient sur l’interdiction des produits phytosanitaires, en la conditionnant

on interdit seulement si on a des alternatives, mais comme vous ne voulez pas ces alternatives, on autorise ! Encore une fois, sous couvert d’arguments économiques et productivistes, la santé des paysans est reléguée au second plan. C’est particulièrement déplorable.

La tendance, que l’on observe depuis quelques semaines, visant à simplifier ou alléger le droit de l’environnement, voire à y déroger, est alarmante. Ce texte s’inscrit pleinement dans ce mouvement d’ensemble. Les offensives contre l’agroécologie relèvent d’une bataille idéologique des rapporteurs : aucune mention du terme dans l’article 1 – pourtant bavard…

Tout au long du texte sont introduits de grands concepts incantatoires qui, au mieux, seront simplement déclaratifs, au pire, constitueront des appuis législatifs pour déroger au respect d’engagements environnementaux. Les articles 13 et 15 – le premier allège le régime de répression des atteintes à la biodiversité, le second accélère les contentieux contre les mégabassines et les fermes gigantesques – sont les deux exemples les plus marquants de ces reculs environnementaux. Je le dis sans concession : ils sont inacceptables. Je suis également inquiet, à un niveau plus global, de la tournure des débats. Outre le fait que nous soutenons deux modèles qui s’opposent, je m’interroge sur le passage en force de certaines dispositions controversées. Le Conseil d’État a par exemple relevé que les notions d’intérêt fondamental de la Nation, d’intérêt général d’intérêt général majeur et de non régression de la souveraineté alimentaire étaient juridiquement floues et donc potentiellement dangereuses. Il a également indiqué que l’article 15 présentait des risques d’inconstitutionnalité. Sur ce même article, la Défenseure des droits a considéré qu’il restreignait « de manière disproportionnée le droit au recours des opposants ». Vous avez fait fi de ces avis, messieurs les rapporteurs, comme vous avez fait fi de la science et des avis de l’Anses et de l’Institut Le texte visait initialement à assurer le renouvellement des générations et à engager l’agriculture sur le chemin des dix prochaines années. En réalité, vous avez profité du contexte pour inclure dans ce projet de loi un panel de mesures érigeant l’agriculture productiviste comme seule et unique méthode, ainsi qu’une succession de reculs environnementaux. De notre côté, à compétitivité et productivité, nous ajoutons revenu agricole juste et respect de l’environnement. Tout cela doit aller de pair ! Le seul modèle viable est celui d’une agriculture raisonnée et à taille humaine, respectueuse des agriculteurs, des consommateurs, de la faune, de la flore et des sols. Pour cela, nous devons en premier lieu assurer aux agriculteurs un revenu juste et rémunérateur. Nous le répéterons jusqu’à ce que nous soyons entendus : nous souhaitons un revenu agricole digne et garanti ! Assurer un revenu juste passe également par une refonte de la PAC pour mettre fin aux inégalités qu’elle entretient de par son mode de distribution. La question du foncier doit également être abordée de la spéculation et du phénomène d’accaparement des terres. Nous devons réguler ! Sans de réelles avancées sur ces thématiques, nous ne redonnerons pas envie et espoir aux générations futures de s’investir dans ce beau métier de paysan. Ces avancées doivent se faire sans renoncer à nos ambitions environnementales et de transition agroécologique. Car il ne faut pas oublier que, sans des sols

sénateurs socialistes, nous ne pouvons pas faire autrement que de voter contre ce texte qui est à des années lumière de proposer des solutions concrètes aux agriculteurs

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après des années d’inaction et d’indifférence face aux souffrances du monde agricole, nous nous réjouissons que cela bouge enfin. La version sénatoriale de ce projet de loi apporte des avancées que nous ne pouvons ignorer. Tout d’abord, nous sommes ravis de voir que sont reprises certaines des propositions que nous portons depuis longtemps comme la priorité aux agriculteurs français, la protection contre la concurrence déloyale ou la lutte contre la surréglementation et l’inflation normative, ce qui marque, pour la première fois depuis bien trop longtemps, une prise de conscience. Le Rassemblement national et Marine Le Pen l’ont toujours affirmé : la souveraineté alimentaire doit être une priorité nationale. On ne vous a pas attendus ! Il était urgent que l’État cesse d’abandonner ceux qui nous nourrissent. Nos agriculteurs n’en peuvent plus. Ils subissent depuis des décennies des politiques qui les étranglent : fiscalité accablante, normes absurdes, distorsions de concurrence insupportables avec des importations qui ne respectent pas nos standards. Pendant que nos paysans se battaient pour survivre, l’État les a trop souvent laissés seuls, prisonniers d’un système qui ne les protège pas. Ce texte apporte enfin une réponse, mais reconnaissons le : ce n’est qu’un début. Ce projet de loi contient des mesures positives. Il amorce une simplification de certaines normes, un allégement partiel des charges et une meilleure prise en compte des contraintes de nos agriculteurs face à la concurrence étrangère. Il prévoit aussi des dispositifs pour mieux structurer les filières et renforcer notre souveraineté alimentaire. Ces avancées vont dans le bon sens, mais elles restent trop limitées pour répondre à l’urgence de la situation. Car la réalité est que ce texte ne s’attaque toujours pas aux racines du problème. Les charges qui pèsent sur nos exploitants restent trop lourdes et les distorsions de concurrence persistent. Nous aurions voulu voir des mécanismes plus contraignants pour interdire l’importation de produits qui ne respectent pas nos normes. Nous aurions voulu une refonte plus ambitieuse de la fiscalité agricole afin de garantir un modèle économique viable à long terme. Nous aurions voulu un cadre plus protecteur pour garantir une juste rémunération aux producteurs. Et vos amis de la Coordination rurale ? Sur tous ces points, ce projet reste encore en deçà des attentes. Nous voterons ce texte, parce qu’il amorce un changement et qu’il serait irresponsable de rejeter ces avancées,

pour veiller à ce que cette première avancée soit non pas un simple effet d’annonce, mais le début d’un véritable renouveau pour notre agriculture. La France ne peut pas être forte et souveraine sans ses paysans. Nous ne laisserons pas leur détresse être de nouveau ignorée ! Mes chers

Si vous disposez d’une délégation de vote, le nom du sénateur pour lequel vous devez voter s’affiche automatiquement sur le terminal en dessous de votre nom. Vous pouvez alors voter pour vous et pour le délégant en sélectionnant le nom correspondant, puis en choisissant une position de vote. Le scrutin est ouvert.

Je voudrais en rappeler quelques points essentiels : notre agriculture élevée au rang d’intérêt général majeur et notre potentiel agricole au rang d’intérêt fondamental pour la Nation les conférences de la souveraineté alimentaire ; la place des femmes en agriculture ; la régénération de l’enseignement agricole ; le diagnostic modulaire pour l’installation ; le droit à l’essai le guichet unique pour accueillir tout projet d’activité agricole ; la dépénalisation des atteintes involontaires et non définitives

des scrutins concernés. J’informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture ainsi qu’à la commission d’enquête sur les pratiques des industriels de l’eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités et la gestion des risques économiques, patrimoniaux, fiscaux, écologiques et sanitaires associés.

visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport, présentée par M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues

contre ceux qui voudraient faire vaciller les valeurs de la République. Après nos écoles, ce sont maintenant nos enceintes sportives qui assistent, impuissantes, aux tentations communautaristes. Je fais ainsi miens les propos du ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, qui déclarait récemment pour lutter contre l’islamisme des Frères musulmans et leur entrisme, il fallait étendre le champ de la laïcité à d’autres espaces publics, par exemple aux compétitions sportives. Si la laïcité garantit la liberté de conscience et la liberté religieuse de chacun, elle pose un cadre à l’exercice desdites libertés : ne pas troubler l’ordre public. Ce postulat fondamental n’étant pas toujours respecté, les acteurs du sport s’accordent sur la nécessité et l’urgence de renforcer certains dispositifs, afin d’assurer à tous une pratique sereine et pacifiée. Concernant l’exercice du sport, depuis de nombreuses années, différents rapports et enquêtes se succèdent pour souligner la fragilité du sport face à la radicalisation et aux dérives contraires aux principes de la République. Pour ma part, j’ai la certitude que les valeurs de dépassement de soi, d’intégration et d’universalité inhérentes au sport permettront d’étendre son accès à tous, quelles que soient l’origine, la religion ou les convictions politiques.

D’aucuns préfèrent se réfugier derrière l’idée selon laquelle ces faits demeurent marginaux. À ceux qui prônent la complaisance face à un phénomène apparemment secondaire, je répondrai d’abord qu’un peu, c’est déjà trop.

s’il est le plus médiatisé, l’exemple des « hijabeuses » n’est que le reflet de revendications qui prolifèrent. Nous le constatons : une question se pose actuellement au sujet du port du voile, qui n’est pas explicitement interdit. Il ouvre à l’émergence de clubs sportifs communautaires promouvant ouvertement le port de signes religieux. Dépassés par les pressions et les menaces dont ils sont l’objet, les dirigeants sportifs, les responsables associatifs et les élus locaux pâtissent d’un flou juridique. ci nourrit confusion et velléités séparatistes en laissant la place aux interprétations divergentes. Notre mobilisation doit être totale pour assurer leur protection.

Cependant, il est regrettable que tous les moyens n’aient pas été mis en œuvre afin d’assurer la neutralité dans la pratique sportive, ce qui provoque régulièrement des incidents ou des dérives. Comme cela nous a été rappelé lors des auditions du rapporteur, certaines fédérations, confrontées à de telles problématiques, se retrouvent démunies face à l’absence de normes strictes et générales édictées par l’État. Si chacun peut, au quotidien et dans le cadre de sa sphère privée, librement pratiquer sa religion, sur un terrain de sport et lors des compétitions, c’est la neutralité qui s’impose. Le Conseil d’État a reconnu aux fédérations sportives délégataires d’un service public la faculté d’interdire, au sein de leurs statuts, les signes religieux ostensibles sur le lieu et pendant la durée des matchs, afin de prévenir tout affrontement ou toute confrontation sans lien avec le sport. Force est de constater que cela ne suffit plus ! Il est donc temps de sanctuariser le domaine sportif, où la neutralité s’impose, et de réaffirmer haut et fort que la République prime la loi religieuse. Il faut donner un vrai soutien législatif aux fédérations. À ceux qui prétendent que ce texte empêcherait certaines femmes de pratiquer une activité sportive, je réponds que les interdictions inscrites dans cette proposition de loi sont strictement limitées aux compétitions sportives organisées par une fédération sportive ayant une délégation de service public.

Cette proposition de loi vise également à donner des moyens législatifs aux élus locaux pour que les équipements sportifs ne soient pas détournés de leur destination. Le service central de renseignement territorial surveille le monde sportif amateur français, où des événements inquiétants se produisent. Une note ainsi des prières sur des terrains de football à Perpignan, le rejet de la mixité dans certains clubs de sport, des pressions exercées sur les encadrants et des éducateurs fichés comme salafistes utilisant des tapis de prière dans les gymnases. Le phénomène découle, selon les auteurs de cette note, d’un repli communautaire observé dans plusieurs quartiers où les fondamentalistes religieux ciblent les jeunes, mêlant sport et pratique religieuse. En particulier, ils transforment les vestiaires et les gymnases en salle de prière. Autre exemple : en novembre dernier, la préfecture de l’Hérault a demandé à la Fédération française de football d’adopter des mesures de suspension à titre conservatoire à l’encontre d’un club en raison de la tenue de rituels de prière accompagnés de musique religieuse, diffusée par les joueurs dans les vestiaires lors de l’avant match.

Les prières au sein des équipements sportifs pendant les entraînements et les compétitions sont incompatibles avec la neutralité exigée par l’État dans le sport. Enfin, il convient également de prévoir dans la loi l’application de la laïcité dans les règlements des piscines. le non respect des règles communes rompt la promesse d’égalité entre les usagers et peut porter atteinte au bon fonctionnement du service public qu’est une piscine municipale. Si certaines actions militantes appellent les femmes à exprimer leurs convictions religieuses au sein des piscines et des espaces de baignade publics, cette vision de la femme et de la liberté d’expression n’est pas celle que reconnaît et promeut la République française. Nous le voyons : ces actions sont délibérément provocatrices. Elles ne visent qu’à diviser, à polariser les opinions et à obliger chacun à prendre parti dans un conflit aux antipodes de la pratique sportive. Face à ces dérives, il est urgent de porter une réglementation claire et ambitieuse dans la loi. Il n’est en effet satisfaisant pour personne que ces questions liées à la pratique religieuse fassent l’objet d’interprétations juridiques différentes selon les lieux et les territoires. il est incompréhensible que le port du burkini soit interdit à Grenoble, mais autorisé à Rennes. L’absence de cadre législatif paralyse la prise de décision, expose les fédérations et limite les moyens de contrôle et les possibilités de sanction du non respect de la neutralité dans le sport. traduit donc l’ambition de nous doter des instruments désormais nécessaires pour lutter contre le communautarisme et le prosélytisme, opérant un juste équilibre entre préservation des libertés individuelles et respect des principes qui unissent la République. Pour défendre les valeurs du sport au quotidien, il faut mener sans faiblesse et sans ambiguïté la lutte contre toute tentative de propagande religieuse ou politique, toute forme de radicalisation religieuse ou de repli communautaire.

la laïcité, l’un des fondements de notre République, inscrite à l’article premier de notre Constitution. La laïcité repose sur un équilibre entre la liberté de conscience dans la sphère privée et la neutralité dans la sphère publique. C’est ce modèle, si singulier à la France, que nous devons préserver, en particulier dans le domaine du sport. En effet, ce dernier est un espace de socialisation et de transmission des valeurs républicaines, un vecteur de l’apprentissage de la citoyenneté au même titre que l’école. Ouvrons les yeux ! Alors que 58 % des licenciés sont âgés de moins de 20 ans, 6,3 millions d’entre eux ayant entre 1 et 13 ans, le sport joue un rôle central dans l’éducation au respect des règles communes et à l’égalité. Les valeurs fondamentales du sport sont des valeurs citoyennes. Les seules règles et les seules différences admissibles sur le terrain sont ainsi celles qu’induit le sport lui même. Nulle stigmatisation ne doit être permise. En particulier, les revendications politiques ou religieuses n’ont pas leur place dans le sport, comme le rappelle le 2 de la règle 50 de la Charte olympique : « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. » Les atteintes à la laïcité dans le sport ne sont pas un phénomène récent, mais elles ont trop longtemps été minimisées, occultées, voire encouragées. Nous ne devons plus renoncer à traiter ce sujet, sans quoi nous risquons le développement rampant d’un communautarisme contraire à nos valeurs. Dès 2003, le rapport de Bernard Stasi sur l’application du principe de laïcité dans la République signalait l’émergence d’équipes qualifiées de « communautaires ». Son auteur regrettait, en outre, le recul de la pratique sportive féminine dans certains quartiers – déjà à l’époque Nous ne pouvons plus accepter cette seule alternative : se soumettre à la nouvelle règle érigée par quelques uns ou s’exclure et laisser le champ libre au communautarisme.

Qualifiée d’inopportune et d’inapplicable à l’époque, cette loi ne souffre plus, aujourd’hui, aucune contestation. Pour paraphraser Jean Zay, selon qui « les écoles doivent rester l’asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas », le sport doit rester la citadelle imprenable sur laquelle les attaques à la laïcité se fracassent. Ainsi, il est le nouveau terrain d’expression de ce que nous appelons aujourd’hui le « séparatisme ». Ce phénomène est désormais largement documenté par plusieurs rapports parlementaires récents, notamment celui de la commission d’enquête du Sénat de 2020 sur la radicalisation islamiste Les atteintes à la laïcité prennent des formes variées et ne sont évidemment pas toutes de même nature. Cependant, elles font l’objet d’un constat partagé par de nombreux acteurs, témoins de la progression inquiétante de comportements remettant en cause le vivre ensemble et l’universalité du sport. Ces atteintes sont, certes, difficiles à quantifier au sein des 360 000 associations sportives, mais quelques chiffres permettent néanmoins d’illustrer le phénomène. cinq ans, 592 alertes ont été rapportées aux cellules de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire

prières collectives dans les vestiaires et sur les terrains, demandes de modification de l’horaire des matchs, rejet de la mixité, ou encore refus de saluer l’adversaire. Les disciplines les plus touchées sont le football, les sports de combat, le tir à l’arc et la musculation. Ces phénomènes sont difficilement quantifiables, mais les occulter serait désormais une faute. Nous ne pouvons pas, en tant qu’élus, rester indifférents aux multiples alertes qui nous sont adressées, lesquelles témoignent d’une érosion progressive du lien social. Dans ce contexte, la proposition de loi de notre collègue Michel Savin est bienvenue. En effet, les outils existants sont insuffisants. Tout d’abord, le contrat d’engagement républicain (CER), introduit par la loi du 24 août 2021, intéressant, mais trop peu mobilisé. Loin d’être un véritable engagement, il est perçu dans les faits comme une simple formalité administrative, sans véritable portée contraignante,

Les services de l’État, notamment les préfectures et les services déconcentrés du ministère chargé des sports, manquent de moyens pour mettre en œuvre efficacement des contrôles, malgré une prise de conscience récente.

de « tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » lors des compétitions. Le Conseil d’État en outre, dans cette même décision, que des limitations à la liberté des licenciés sont possibles « si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Par ailleurs, dans une ordonnance du 21 juin 2022, le Conseil d’État a validé la suspension par le représentant de l’État du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble, qui autorisait alors le port du burkini. Ces décisions ont encouragé plusieurs fédérations à adopter des règlements interdisant le port ostensible de signes religieux ou politiques en compétition, notamment les fédérations françaises de football, de basketball et de volleyball. D’autres n’ont pas encore statué, mais des pressions s’exercent sur elles. Il est donc temps de fixer un cadre juridique commun qui protège l’ensemble des fédérations sportives. La cohérence globale du message que le législateur doit émettre est essentielle pour mettre fin à la confusion largement exploitée par ceux qui veulent détruire notre modèle républicain. franciliens de basket ont adressé l’an dernier une pétition à la Fédération française de basketball à la suite de l’interdiction, par celle ci, du « port de tout équipement à connotation religieuse ou politique ». Des campagnes sont également relayées sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, en effet, si les fédérations sportives ont la faculté de mettre en place des limitations, elles n’en ont pas l’obligation, ce qui crée la confusion. Rien ne peut justifier qu’un principe aussi fondamental que celui de la laïcité s’applique différemment d’une discipline à l’autre.

prévoit l’interdiction de tout exercice d’un culte dans les locaux mis à disposition par les collectivités territoriales en vue d’une pratique sportive, afin de ne pas dévoyer leur usage. il a pour objet de faire respecter les mêmes principes de neutralité et de laïcité dans les piscines et les espaces de baignade artificiels publics. En commission, nous avons complété le texte afin de permettre

auprès du ministre de l’intérieur,

L’été dernier, notre pays a accueilli les trente troisièmes Jeux de l’ère moderne. Le succès des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a transcendé tous les courants de pensée, les identités singulières et les particularismes. Nous avons su faire nation.

Les salles et les terrains de sport ne peuvent en aucun cas devenir de nouveaux espaces d’expression du séparatisme. Il nous faut réaffirmer notre conviction

discours se réclamant des droits fondamentaux et des libertés individuelles pour faire progresser un agenda séparatiste. Tel était bien l’objectif véritable des « hijabeuses » lorsqu’elles ont brandi le principe de non discrimination pour s’affranchir des règles communes. C’est d’ailleurs le principe même de l’entrisme : faire reculer, étape par étape, petit à petit, les garde fous de l’universalisme pour installer peu à peu une société communautarisée et divisée, une société dont nous ne voulons pas.

Depuis quelques années, nous avons d’ailleurs renforcé notre arsenal législatif, nous dotant d’instruments utiles pour défendre partout les valeurs de notre République. Le vote de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a constitué un moment important de cette stratégie qui se veut globale.

possible. À l’article 1, l’amendement n° 31 vise à préciser que l’interdiction du port de tout signe religieux ostentatoire s’applique aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires de service public. C’est en effet au nom du service public que le principe de laïcité s’impose.

Il ajoutait même : « Ma position est très claire, pas de religion dans les clubs et l’État ne reconnaîtra pas et ne versera pas un centime à ceux qui sortent du cadre. »

Cette vision, inspirée d’un célèbre slogan publicitaire – « Venez comme vous êtes » –, interroge sur l’application du principe de laïcité dans le cadre sportif. Le premier alinéa de l’article premier de la Constitution de 1958 dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale

Notre responsabilité collective est de sécuriser le sport, cet espace partagé de dépassement et d’éducation aux valeurs de la République, en appliquant des règles communes de pratique.

ou de handball, par exemple, alors qu’elles pratiquent la même activité au collège ou au lycée sans signe religieux ? J’estime que non. Peut on se contenter de constater que les infrastructures sportives mises à la disposition des clubs par les collectivités locales soient transformées en lieux de prière ? La réponse est encore non.

d’interprétations susceptibles de fragiliser les règles de la République. En tant que sénateur, mais aussi en tant que professeur de judo, je me réjouis que cette proposition de loi permette la mise en place d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des éducateurs sportifs n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Il est essentiel d’empêcher ces professionnels, dont certains font l’objet d’un suivi par les services de renseignement, d’utiliser le sport comme un vecteur de prosélytisme auprès de nos enfants et de nos jeunes. Enfin, l’article 3 apporte une réponse législative à la compromission, ou peut être seulement à la faiblesse de certains élus face à l’islamisme radical, en imposant l’inscription, dans les règlements intérieurs des espaces de baignade, de l’interdiction de tenues aquatiques à caractère religieux. Le fait qu’un maire autorise le port d’une tenue à caractère religieux dans une piscine municipale constitue une rupture manifeste de l’égalité de traitement des usagers, susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public et, par

les collectivités territoriales, les élus, les fédérations, les associations de toute forme de prosélytisme idéologique ou religieux. Je vous invite donc à soutenir ce texte,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui d’une proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le domaine du sport.

nous émettons quelques réserves sur la rédaction actuelle de ce texte. Notre système républicain repose sur un principe de laïcité qui garantit à chacun la liberté de conscience, dont découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions

du risque d’un trouble à l’ordre public. Le principe de neutralité ne s’appliquant qu’aux activités sportives organisées par les collectivités publiques ou les fédérations sportives agréées chargées d’une mission de service public, le champ du dispositif paraît

sa décision du 29 juin 2023, confirmant la possibilité, pour la Fédération française de football, de prévoir dans ses statuts, dans le cadre de sa délégation de service public et pour le bon déroulement des compétitions et manifestations qu’elle organise ou autorise, l’interdiction du port

Au même titre que l’école, le sport initie en effet nos enfants à la coopération et au respect des règles communes. Il est un facteur d’intégration, de mixité sociale et de renforcement de la cohésion nationale. Au nom de mon groupe, je proposerai donc de circonscrire l’application du dispositif proposé par cette

Une fois amendé comme nous l’espérons, ce texte constituera un levier de protection des droits de chacun dans le respect d’un cadre républicain, mes chers collègues. Il permettra aux jeunes de grandir et d’évoluer dans un environnement sportif respectueux et libre de toute pression religieuse.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe RDSE, par son histoire et sa philosophie, se réjouit toujours de l’attention portée à la laïcité. nous avons trop souvent négligé cette dernière. André Comte Sponville définit la laïcité comme « une volonté : celle de vivre ensemble, pacifiquement et librement, quelle que soit la religion ou l’irréligion des uns et des autres

un vecteur d’apprentissage des valeurs de respect et de fraternité. Elle doit être encouragée pour tous. Que doit être la laïcité dans le sport ? Avant tout, le respect de celui qui croit et de celui qui ne croit pas. Cette proposition de loi a un objectif essentiel, celui de protéger la laïcité. Dans sa rédaction actuelle, elle risque toutefois de restreindre indûment certaines libertés individuelles.

L’article 1 de ce texte généralise l’interdiction, déjà prévue par certaines fédérations, du port de signes religieux ostensibles durant les compétitions.

sportive. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire peut déjà autoriser ou interdire un rassemblement religieux dans un lieu public si ce rassemblement contrevient à la tranquillité, la salubrité, la sécurité ou le bon ordre public.

L’article 3 impose le respect des principes de neutralité et de laïcité dans les piscines et les espaces de baignade artificiels publics, notamment par l’interdiction du port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse.

légitime. Cette proposition de loi vise à protéger le sport, vecteur d’apprentissage de la citoyenneté, des atteintes à la laïcité. Des acteurs de terrain évoquent l’accroissement du nombre de telles atteintes, qui relèveraient d’un repli communautaire.

que celui, non moins excellent, de notre rapporteur Stéphane Piednoir. La laïcité est l’un des piliers de notre République. Elle garantit la neutralité de l’État et assure l’égalité de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances. Garantir l’égalité de traitement des usagers dans l’espace sportif est essentiel pour préserver la cohésion sociale et éviter toute forme de discrimination.

Ces données illustrent la réalité et l’ampleur des défis que nous devons relever, mes chers collègues. Il faut bien comprendre que la laïcité vise non pas à exclure, mais à protéger. Très bien ! Elle garantit que chacun puisse pratiquer son sport librement, sans subir de pression religieuse ou communautaire.

En tout état de cause, le sport doit rester un lieu de rencontre et de partage, au delà des différences individuelles. Force est pourtant de constater que nous ne sommes plus en mesure de compter les atteintes à notre principe de laïcité. Les incidents observés, notamment les annulations de match, montrent la nécessité de règles claires et uniformes pour préserver la paix sociale et l’union nationale. Certains promoteurs d’une vision radicale et politique de la religion tentent du reste d’imposer des pratiques incompatibles avec notre société. Cette proposition de loi permettra de sécuriser le respect du principe de laïcité lors des manifestations sportives.

qui donne aux fédérations sportives la possibilité de prendre des mesures limitant la liberté d’expression et de conviction afin de garantir « le bon fonctionnement du service public [et] la protection des droits et libertés d’autrui ». Nous ne comptons plus les incidents qui se sont déroulés dans des stades à cause du port de tenues ou de signes religieux. Plusieurs fédérations, notamment la Fédération française de football

sportive. Cette mesure va dans le bon sens, car elle permettra à chacun de pratiquer un sport, quelle que soit son appartenance religieuse. Le principe de laïcité doit s’appliquer dans les locaux publics.

Il ne faut d’ailleurs pas se cacher derrière un éventuel trouble à la salubrité publique ou derrière un motif d’hygiène pour interdire le port des vêtements religieux : nous n’avons pas besoin de prétexte. Nous sommes dans une République laïque. C’est ce principe qui doit prévaloir.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Charte olympique du Comité international olympique (CIO), dans sa version en vigueur au 30 janvier 2025, reconnaît comme principes fondamentaux de l’olympisme le droit de pratiquer un sport sans discrimination, la neutralité politique des compétitions et la liberté d’expression de leurs participants. En outre, sa règle 50.2 stipule : « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Cette interdiction est la condition d’observation des principes fondamentaux cités à l’instant. C’est parce que les compétitions sont neutres que leurs participants ne subissent aucune discrimination et que leur liberté d’expression est protégée. telle logique n’est pas sans rappeler celle de la laïcité française, qui garantit la liberté de conscience des individus en exigeant de l’État qu’il ne reconnaisse aucun culte. La neutralité est une condition de cette liberté. Certes, la loi de 1905 ne l’impose pas aux usagers des services publics, seuls leurs agents y sont soumis, mais l’athlète qui participe à une compétition n’est pas un simple usager. L’essence de l’éthique olympique est d’organiser des compétitions entre des athlètes placés sur un pied d’égalité. Ces derniers ne confrontent que leur force, leur adresse, leur intelligence et leur esprit d’équipe, en dehors de toute autre considération étrangère au sport. En cela, l’olympisme organise un espace universel par une langue commune fondée sur les seules règles sportives. Alors que, partout sur la planète, l’universalisme est battu en brèche par les particularismes religieux, les revendications identitaires ou politiques, il appartient à la France à la France de le protéger, parce qu’elle a activement participé à la construction de l’olympisme depuis son premier congrès, tenu à la Sorbonne en 1894. Il nous appartient de surcroît de défendre l’esprit de la contre les instances chargées de l’appliquer : je regrette vivement que le CIO et certaines fédérations internationales aient accepté des transgressions de la règle commune pour satisfaire des États qui interdisent aux femmes de choisir librement ce qu’elles doivent porter. Ces violations de la Charte olympique fragilisent le combat des femmes qui s’en réclament pour se défendre. chers collègues, quelle est la liberté d’une athlète iranienne de ne pas porter une tenue religieuse, si l’application du principe de neutralité olympique est laissée à la seule appréciation des délégations ?

Hassiba Boulmerka, médaillée d’or en 1992, et de la Tunisienne Habiba Ghribi, médaillée d’or en 2012. Toutes trois ont refusé la tenue religieuse que les hommes voulaient leur imposer. Pour défendre leur liberté, il nous faut défendre la Charte olympique. L’introduction dans le droit français de l’obligation de neutralité pour les compétitions, telle qu’elle est édictée par l’article 50.2 de la Charte olympique, aurait été une façon de la promouvoir au sein des instances internationales. Cela aurait de protéger les fédérations françaises qui l’ont reprise dans leur règlement et qui sont aujourd’hui soumises aux pressions de ceux pour qui l’impératif religieux doit primer la loi commune. Je regrette donc que la rédaction de l’article 1 du présent texte ne s’en éloigne, en ne retenant que « le port de signes ou de tenues », alors que la Charte olympique proscrit les « démonstrations », ce qui inclut les gestes, par exemple les saluts nazis. De manière plus générale, cette proposition de loi a heureusement suscité une réflexion utile quant à la nécessité de préciser la nature des missions de service public confiées par l’État aux fédérations sportives. Parce qu’elles accueillent de nombreux mineurs, les fédérations participent au service public pour l’éducation de la jeunesse par le sport.

il vous appartiendra de lancer cette réflexion pour que l’héritage des jeux Olympiques soit non seulement matériel, mais aussi moral et législatif. La parole est

Jean Jaurès, n’est autre chose que l’égalité des droits. Or il n’y a pas égalité des droits si l’attachement de tel ou tel citoyen à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause de disgrâce. »

vous visez directement, frontalement et lâchement, des femmes de confession musulmane de notre pays. Voilà la réalité : nous examinons un texte cherchant à exclure les musulmans.

J’étais prise au piège entre ma passion [pour le football] et quelque chose qui constitue une très grande partie de mon identité. C’est comme si on avait essayé de me demander de choisir entre les deux. Hélène : « Je suis allée à des matchs, parfois j’ai décidé de ne pas y aller parce que c’était trop difficile et je n’avais pas la force d’encourager mes coéquipières. Cela change la manière dont je m’entraîne, car je vais aux entraînements pour m’amuser maintenant, mais aussi pour progresser individuellement ; et c’est dur de progresser individuellement si on ne peut pas jouer pendant les matchs, c’est dur de rester motivée sans les matchs. « Je suis une joueuse compétitive, je ne vais pas mentir. Je l’ai toujours été, depuis l’âge de 5 ans. Donc c’est un élément essentiel de votre passion dont on vous prive, même physiquement, parce que les entraînements sont souvent moins intenses que les matchs. Mentalement, c’est difficile aussi, parce qu’on se sent vraiment exclue. Tout le monde sait pourquoi vous ne jouez pas ; surtout si vous allez vers le banc et que l’arbitre vous dit d’aller dans les gradins, tout le monde vous voit aller du banc aux gradins. » Rien ne l’empêche de jouer ! « Pour le reste du monde, c’est juste une question de ne pas pouvoir jouer, mais pour vous c’est une marche de la honte. Assma : « Ça m’impacte beaucoup. Mais je veux continuer à me battre, vraiment. Je veux continuer à me battre, parce que par exemple ce sport, le volleyball, ça m’a beaucoup, beaucoup aidée dans le rapport au corps que j’avais. On dit souvent : “le sport, c’est un vecteur d’émancipation”.

Le sport est le terrain de la solidarité et de la cohésion : nous refusons qu’il devienne celui de la discrimination. Eh bien… Le 28 octobre dernier, trois rapporteurs spéciaux de l’ONU et le groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles ont d’ailleurs estimé que l’interdiction du couvre chef,

Une laïcité éclairée, qui protège la liberté de conscience et la neutralité de l’État, ou une laïcité instrumentalisée à des fins identitaires et partisanes ? Mes chers collègues, ce débat n’est pas qu’une affaire de règlements ou de codes. Il met en jeu notre pacte républicain et la manière dont nous concevons le vivre ensemble. La laïcité n’est pas une arme,

par cette proposition de loi d’interdiction, faire de la laïcité un outil d’exclusion, c’est travestir son essence. User d’elle comme d’un prétexte pour dicter aux individus ce qu’ils doivent être, c’est détourner un principe de notre République au profit d’une lecture restrictive

Dans cet esprit, je me permets de vous rappeler que les garanties constitutionnelles interdisent non seulement de cibler une religion plus qu’une autre, mais aussi de porter une atteinte excessive et disproportionnée aux libertés individuelles. Force est de constater que, depuis plusieurs années, la droite ne cesse d’interroger notre manière de vivre ensemble. Alors, reprenons le débat. Confrontons votre vision étriquée de la laïcité à la nôtre

En interdisant de manière générale l’utilisation d’un équipement sportif comme salle de prière, il va à l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’État et de l’esprit même de la loi de 1905, qui autorisent sous condition la mise à disposition temporaire de locaux communaux à des associations cultuelles. Vous le savez bien. Nous prenons acte de l’amendement de M. le rapporteur

Deuxièmement, cette proposition de loi est discriminatoire. En ciblant spécifiquement les signes religieux, notamment le voile, elle marginalise en particulier nos concitoyennes musulmanes, trop souvent au centre des polémiques relatives De telles interdictions entraîneront à coup sûr une exclusion sociale dévastatrice pour ces femmes, pour qui le sport est un canal essentiel de sociabilité, d’intégration et de bien être physique et mental.

de loi interdit, lors des compétitions, « le port de tout signe ou tenue manifestant [clairement] une appartenance politique ou religieuse ». Dès lors, je m’interroge : la majorité sénatoriale entend elle aussi interdire les campagnes contre l’homophobie, qui se manifestent parfois par le port d’un autocollant sur le maillot pendant les matchs ? Voyez, chers collègues de droite, à quoi vos amalgames pourraient mener… Troisièmement, cette proposition de loi est potentiellement liberticide. Elle permet de restreindre les libertés individuelles sans fournir de justification suffisante, pavant ainsi la voie à des interprétations dangereuses, car extrêmes, de la laïcité. Le Conseil d’État lui même a souligné que de telles mesures généralisatrices n’étaient ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées. Cette proposition de loi constitue une violation flagrante des engagements internationaux de la France en matière de droits humains. Elle va à l’encontre de tout ce que notre République représente. Afin de préserver l’attractivité de la France pour l’accueil d’événements sportifs internationaux, cette nouvelle réglementation, si elle était adoptée, ne s’appliquerait pas aux compétitions inscrites au calendrier des fédérations internationales.

Tout simplement le sport, dans son essence la plus pure. Vecteur d’intégration et de cohésion sociale, le sport est un domaine où les différences de foi, de couleur ou de conviction s’effacent devant le mérite, l’effort et le respect mutuel.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand Karim Benzema et de nombreux autres footballeurs professionnels français « aiment » le post Instagram d’une célébrité tchétchène célébrant la décapitation de Samuel Paty, c’est qu’il y a une emprise islamiste au plus haut sommet du sport français. La défaite du football français, qui avait commencé par des accommodements raisonnables sur les repas halal des joueurs, finit avec l’apologie du terrorisme. Voilà où mène notre lâcheté face à la pernicieuse politique des petits pas menée par les Frères musulmans, accompagnée des grands pas de la gauche… La soumission islamiste commence toujours par la victimisation. Elle se poursuit par la revendication, puis elle s’impose par l’intimidation.

En 2025, en France, des clubs de football professionnels se soumettent à la charia, en diffusant des photos de leurs joueurs masculins genoux floutés, selon les codes de la pudeur islamique.

Leur objectif est de nous asservir à leur code religieux, qui, rappelons le, est aussi un code civil. Aujourd’hui, le législateur français doit faire barrage pour protéger les présidents de fédération sportive, les présidents de club et les 16,5 millions de nos compatriotes licenciés d’une fédération sportive, pris en otages par un entrisme islamiste victimaire, organisé et menaçant. La parenthèse enchantée des jeux Olympiques et Paralympiques cache les petits maîtres chanteurs de l’islamisme, qui marquent leur terrain au quotidien dans les clubs de banlieue ou de province.

Nous avons tous en tête le soutien du maire islamo écolo collabo de Grenoble, jamais en retard d’une régression, qui a soutenu l’association des « hijabeuses comme il voudrait imposer des créneaux pour les burkinis dans ses piscines municipales. Ces élus prennent pour mot d’ordre « vivre le sport ensemble » ; mais ils font advenir l’apartheid, la discrimination à l’égard des femmes et le face à face. Même les plus hautes institutions ont capitulé. L’art de la nuance… En effet, la sentence « la liberté est dans le hijab » ne vient pas de Téhéran, mais d’une campagne de promotion concoctée par le Conseil de l’Europe à Bruxelles. Face à cela, face à ces collabos, la France ne doit rien céder.

après midi un texte majeur, qu’il s’agisse des valeurs de la République ou de la lutte contre le communautarisme. Face à la multiplication des phénomènes de repli communautaire dans le sport, aucun renoncement n’est acceptable. Il est de notre devoir d’agir en responsabilité. Il y a déjà plus de vingt ans, le rapport de la commission Bernard Stasi sur l’application de la laïcité alertait quant à la formation d’équipes « communautaires » et quant au déclin de la pratique sportive féminine.

les fédérations sportives sont confrontées à des revendications communautaires croissantes. Face à cela, le renoncement n’est pas une option.

Cette levée de boucliers doit se poursuivre et s’intensifier, car le repli communautaire et le séparatisme n’auront jamais leur place dans le sport. Fondateur des jeux Olympiques modernes, Pierre de Coubertin disait du sport qu’il faisait « partie du patrimoine de tout homme et de toute femme », et que rien ne pourrait jamais « compenser son absence Le sport a le pouvoir de rassembler des Français de toutes origines sociales, culturelles et territoriales. Il est, en ce sens, un puissant vecteur d’intégration et de cohésion.

titre, l’interdiction du port de signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives, édictée à l’article 1, est essentielle. Parmi les phénomènes de repli l’un des plus récurrents et des plus largement rejetés par la société française est évidemment le port de signes religieux visibles. Il en va de même de l’interdiction des prières collectives dans les locaux mis à disposition par les collectivités territoriales en vue d’une pratique sportive, ainsi que du respect des principes de laïcité et de neutralité dans les piscines publiques, conformément aux articles 2 et 3. Le présent texte permet également la réalisation d’enquêtes administratives préalables à la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif. Cette disposition est d’autant plus urgente que, en l’état actuel du droit, un individu fiché au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste peut tout de même se voir délivrer une carte professionnelle d’éducateur sportif.

Ce n’est ni plus ni moins qu’un renoncement. Cette posture revient à admettre dans le sport la discrimination de genre que certaines religions imposent aux femmes et à nier que le port de vêtements religieux peut représenter une pression pour les autres femmes de même confession. En quoi le fait d’autoriser le port du voile lors d’activités sportives permettrait il d’émanciper, d’intégrer et d’assimiler de jeunes femmes ? En rien ! Exactement ! On ne répond pas aux prédicateurs et à ceux qui dévoient le sport pour y faire du prosélytisme par le renoncement. Or refuser de faire respecter la laïcité dans le sport, au motif que cela éloignerait certaines femmes, c’est, je le La meilleure façon de défendre les femmes, le sport et la laïcité, c’est de respecter nous mêmes nos propres valeurs, d’être fidèles à nos principes et de refuser toute compromission. C’est pourquoi le groupe Les Indépendants soutient les objectifs de cette proposition de loi. Oui, la laïcité doit être protégée

pourquoi est il urgent de légiférer pour assurer le respect du principe de laïcité dans le sport, et ce dans un pays dont la Constitution dispose clairement, dans son article premier, qu’il « est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »

Gabriel Attal, lors de son passage au ministère de l’éducation nationale, avait tenu un discours ferme vis à vis de l’entrisme religieux à l’école. Nous demandons à Mme la ministre des sports de faire preuve de la même fermeté au sein de son ministère. Le voile, l’abaya, le qamis, le burkini ne sont pas des vêtements culturels, ce sont des étendards politiques qui s’immiscent dans notre société et, tout particulièrement, dans le sport.

Le port de l’abaya par de plus en plus de petites filles en est un exemple effrayant qui, en France comme ailleurs, contribue à un véritable apartheid sexuel. N’oublions pas qu’en Iran le premier geste politique des mollahs, à leur arrivée au pouvoir en 1979, a consisté à voiler les femmes et à les rendre invisibles, alors que ce pays était jusqu’alors très moderne et à l’avant garde du féminisme. N’oublions pas non plus

a ainsi foulé aux pieds l’article 50 de la Charte olympique. C’est dans ce même pays que des femmes meurent aujourd’hui, parce qu’elles refusent de porter ce voile qui étouffe leur cri : « Femme, Vie, Liberté ». Le sport fait fi de la religion, du milieu social, de la couleur de peau et permet de se réunir sous un même maillot, avec un même objectif : gagner, battre l’adversaire. Cette saine émulation est une chance, en particulier pour la jeunesse. Sachons absolument la préserver, tout comme il faut rappeler que les équipements sportifs ne sont pas destinés à se transformer en lieux de culte. Bravo ! Une fois n’est pas coutume, je vais citer le Président de la République, discours des Mureaux en octobre 2020, avait déclaré : « Ce à quoi nous devons nous attaquer, c’est le séparatisme islamiste. C’est un projet conscient, théorisé, politico religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, […] dont les manifestations sont […] le développement de pratiques sportives, culturelles communautarisées qui sont le prétexte pour l’enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C’est l’endoctrinement et par celui ci, la négation de nos principes, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. » Plus de quatre ans

Pour conserver ses vertus émancipatrices et libératrices, pour les jeunes et les moins jeunes, le sport doit se pratiquer sans entrave religieuse. Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir l’hydre islamiste

notre rôle est d’affirmer que la neutralité dans le sport répond à une impérieuse nécessité. Ne soyons pas dupes, ne nous voilons pas la face, le sport fait partie des vecteurs de l’entrisme islamiste, vecteur déjà préconisé par le fondateur des Frères musulmans, Hassan el Benna, décédé en 1949, dont je rapporte ici les propos Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. » Monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’écrivait Pierre de Coubertin, il est temps, dans le domaine du sport comme dans tous les autres, de « voir loin, parler franc, agir ferme

Mais l’essence même du sport, aujourd’hui comme demain, et si nous y veillons, réside dans sa capacité à rassembler, à unir autour d’une même passion des femmes et des hommes venus d’horizons variés. Dans une société de plus en plus archipélisée, bunkérisée, « escargotisée », le rectangle vert, le stade et le vestiaire sont parmi les derniers espaces de mixité sociale. Combien de membres d’une même association sportive, issus néanmoins de milieux différents, ne se seraient peut être jamais rencontrés sans le sport ? Quand on porte le même maillot, les chaînes religieuses, les de classe, les stigmates des quartiers s’effacent. sous un même maillot, plus de barrières, que des coéquipiers ! Quand on joue ensemble, quand on souffre ensemble, quand on gagne et qu’on perd ensemble, on apprend à se connaître, à s’apprécier, à se comprendre. Le vestiaire peut être cet endroit où tombent les préjugés et où naît la fraternité. Faire partie d’une équipe est un formidable moyen d’intégration et de cohésion sociale. Les clubs sportifs demeurent d’incomparables lieux d’échanges, d’amitié, de générosité, où la formule latine – « un esprit sain dans un corps sain » – prend tout son sens pour le bien de tous. Le sport ne divise pas, il rassemble. Quand l’essentiel, c’est l’équipe, les différences s’estompent. Que la religion reste donc aux portes du stade et du gymnase, il y a assez de facteurs de division dans notre société ! La parole est à M. Jean

nous entendons défendre cette position dans tous les domaines de la vie publique et non simplement dans le sport. Car on pourrait très bien légiférer demain sur d’autres secteurs de la vie associative que le secteur sportif.

de la réponse apportée entre ces différents risques et le respect des libertés constitutionnelles d’expression, de pensée et d’exercice de sa religion. La loi de 1905 et la jurisprudence du Conseil d’État sont extrêmement claires. La dérogation introduite par la loi de 2004 pour les élèves de notre pays, catégorie d’usagers particulière, extrêmement influençables du fait de leur âge, est amplement suffisante. Nous

principalement au niveau amateur. Nous défendons encore et toujours une vision fidèle aux principes fondamentaux de notre République et, plus particulièrement, à l’esprit de la loi de 1905. Cette loi, qui régit la séparation des Églises et de l’État, impose un principe de neutralité aux agents du service public et non à ses usagers. Il s’agit d’un principe constant et clair, confirmé à maintes reprises par le juge administratif. En réalité, l’interdiction absolue du port de signes religieux dans le sport ne résoudrait aucun problème ; elle en créerait même de nouveaux. Elle alimenterait la stigmatisation et les tensions au lieu de favoriser un climat de respect et de tolérance. Le sport ne doit pas exclure. Fidèles à notre engagement en faveur des libertés individuelles et du vivre ensemble, nous demandons la suppression de cet article.

Pourquoi mettre sur le même plan le sport et l’école ? C’est parce que toutes les auditions que nous avons menées confirment que ce sont les deux vecteurs principaux de séparatisme. Madame Ollivier, j’étais enseignant en 2004,

par ailleurs que le Conseil d’État a estimé que les fédérations sportives étaient chargées d’assurer le bon fonctionnement du service public, dont la gestion leur est confiée, et peuvent à ce titre imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues lors des compétitions et manifestations sportives. Enfin, comme

Je vous rappelle que cette loi a été prise sur le fondement de la liberté de conscience, non pas pour neutraliser l’école, mais pour protéger la liberté de conscience de jeunes esprits en

en dehors des règles religieuses. Pour l’instant ! La laïcité est une chance pour tous les jeunes Français, pour toutes les femmes françaises et j’ai une pensée pour les femmes qui luttent et prennent des coups tous les jours dans les quartiers, parce qu’elles ne veulent pas subir ces pressions islamistes

! Si une femme veut porter un signe religieux lors d’une compétition sportive, c’est qu’elle met la religion au dessus de ces règles. Sérieusement

de loi permettra tout simplement de dépassionner le débat et même de le faire disparaître : vous verrez,

presse : « Réduire la question de l’islam – puisque c’est votre obsession, mes chers collègues – à un phénomène d’islamisme ou d’islamisation est très mal à propos. Il n’y a pas, je le redis, une volonté de conquête de l’espace.

que la conséquence d’une politique d’immigration massive, incontrôlée, qui conduit une partie de la jeunesse de France à se reconnaître davantage dans la religion musulmane que dans notre modèle républicain ! La

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

la police des vêtements. L’article L. 100 1 du code du sport garantit un accès libre et sans discrimination aux pratiques sportives. La Constitution proclame l’égalité

Au delà du droit, pensons aux conséquences concrètes, puisque ce texte ne protégera personne ni ne réglera aucun problème. En revanche, il privera certaines femmes de l’accès au sport de haut niveau, les empêchant de concourir sous le prétexte de leur tenue vestimentaire. Or le sport n’est pas seulement un loisir, c’est aussi un vecteur d’émancipation, d’inclusion et d’égalité.

sans discrimination. Nous établissons donc un délit d’entrave à l’accès au sport, sanctionné par les peines habituelles pour discrimination, afin d’empêcher toute exclusion arbitraire et de garantir l’effectivité du droit de chacun à pratiquer librement le sport.

de trouble à l’ordre public. Nous proposons donc de codifier l’équilibre dégagé par le Conseil d’État dans son arrêt du 29 juin 2023. Le second est de protéger nos enfants. En France, 6,3 millions d’enfants de moins de 13 ans sont licenciés d’une fédération sportive et 58 % des sportifs licenciés ont moins de 20 ans. Au même titre que l’école, le sport initie nos enfants à la coopération et au respect de la règle commune. Il est un facteur d’intégration, de mixité sociale et de renforcement de la cohésion nationale.

En effet, nos enfants, sur le modèle de notre école républicaine, ne doivent pas être influencés dans leurs choix avant leur majorité. Quel est l’avis de la commission

rien au fond. Certes, seules les fédérations délégataires d’une mission de service public, et non toutes les fédérations agréées, devront, comme leurs organes déconcentrés, les ligues et les clubs, interdire le port ostensible de signes religieux et politiques durant les compétitions départementales, régionales et nationales.

Je comprends l’appel à la vigilance de Michel Savin, mais je trouve l’amendement du Gouvernement intéressant. Remontons le temps pour faire un peu d’histoire. La laïcité, c’est d’abord la neutralité des agents du service public.

Le constat est simple. Aujourd’hui, de nombreuses fédérations sportives disposent déjà dans leur règlement de sanctions disciplinaires en cas de non respect du principe de laïcité. C’est notamment le cas de la fédération française de football. football. Nous proposons de généraliser et d’harmoniser cette pratique en prévoyant explicitement que toute violation du principe de laïcité sera sanctionnée selon les règles disciplinaires propres à chaque fédération agréée et à chaque ligue professionnelle. Il s’agit non pas de créer de nouvelles sanctions, mais bien de donner une base légale claire aux dispositifs existants tout en respectant l’autonomie des fédérations dans la définition de leur échelle de sanctions. Cette approche pragmatique permettra de garantir que le sport, vecteur essentiel de cohésion sociale dans notre République, demeure cet espace de neutralité

Mme Else Joseph. Les grandes manifestations sportives témoignent depuis toujours du rôle central du sport comme vecteur de cohésion sociale. Elles constituent un précieux moment d’unité nationale et ne sauraient être ternies par des considérations politiques ou religieuses. Étrenner le maillot français, c’est porter ses valeurs valeurs ! La loi confie l’exécution d’un service public aux fédérations sportives, tenues d’assurer l’égalité des usagers et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité. Ces fédérations exercent un pouvoir de direction sur les sportifs arborant le maillot de l’équipe de France, qui participent dès lors à une mission de service public. À ce titre, ils doivent être soumis au principe de neutralité. C’est ce que le Conseil d’État a expressément reconnu par un arrêt du 29 juin 2023. Lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Gouvernement a également réaffirmé que la neutralité s’imposait à ces athlètes. Aujourd’hui, si cette nécessité est assez communément admise, aucune loi n’impose clairement la neutralité aux personnes sélectionnées en équipe de France. C’est dans ce flou juridique que s’engouffrent les revendications communautaristes de celles et de ceux qui voudraient faire vaciller les valeurs de la République française. inscrire dans le droit que le principe de neutralité s’applique aux personnes sélectionnées en équipe de France, afin de veiller au respect du principe de laïcité et de protéger les fédérations face aux tentatives de dévoiement communautaires.

qui les a sélectionnés. C’est à ce titre qu’ils doivent respecter le principe de neutralité que vous évoquez. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs confirmé dans sa décision du 29 juin 2023.

le dispositif envisagé par l’auteur de la proposition de loi, en étendant son application aux athlètes français sélectionnés par les fédérations délégataires de services publics. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable

Toutefois, il est primordial que ces règles soient adoptées en parfaite connaissance du cadre juridique et des principes fondamentaux de notre République, notamment en matière de laïcité et de lutte contre les discriminations. même la laïcité est dénaturée et instrumentalisée, alors s’impose la nécessité de clarifier l’application de ce principe dans le sport. Il est indispensable de former les instances dirigeantes, notamment en les sensibilisant aux discriminations, directes et indirectes. l’avis de la commission

je suis un peu réservé quant à la rédaction de l’amendement, qui vise à établir un lien entre la laïcité et la notion de discrimination indirecte, ce qui laisse entendre que l’application du principe de laïcité pourrait conduire à des formes insidieuses de discrimination.

champ du sport, qui vise à accompagner les fédérations, a été actualisé et transmis à ces dernières. Il rappelle avec pédagogie, au travers de différentes mises en situation, le périmètre d’application du principe de laïcité. Les contrats de délégation des fédérations mentionnent expressément la lutte contre le séparatisme comme une priorité d’engagement à structurer autour des cadres d’État. Le déploiement de ces référents est en cours. Il revient aux fédérations et aux instances dirigeantes

souhaite revenir sur l’interrogation du rapporteur au sujet du lien entre laïcité et discrimination indirecte. En échangeant avec un certain nombre d’acteurs et d’actrices,

évaluant les conséquences réelles de l’interdiction du port de signes religieux dans les compétitions sportives. Avant d’imposer une telle mesure, il est essentiel de penser aux premières personnes du fait qu’elle constitue un dévoiement de la laïcité, risque d’avoir des effets négatifs, notamment pour les femmes et les jeunes filles, qui rencontrent déjà de nombreuses difficultés pour accéder au sport. Les données sont sans appel 49 % des femmes renoncent à la pratique sportive pour des raisons financières, 46 % en raison de contraintes familiales et 40 % à cause de charges domestiques. Face à ces inégalités persistantes, il est absurde d’ajouter une nouvelle barrière en interdisant à certaines femmes de pratiquer en raison de leur tenue

À l’heure où les femmes sont sous représentées dans le sport, notre priorité devrait être de corriger cette inégalité et de favoriser l’accès des femmes au sport. Or cette proposition de loi pourrait justement avoir l’effet inverse. Elle risque en particulier d’exclure les femmes portant le voile de la pratique sportive. C’est une inquiétude qui est largement partagée.

L’arrêt du sport chez les adolescentes est par ailleurs un phénomène massif et préoccupant. Selon un rapport de l’Unesco de 2024, une fille sur deux arrête le sport à l’adolescence. Or cette sédentarité entraîne de lourdes conséquences sur leur santé physique et mentale. Puisque le sport a vocation à être un vecteur d’émancipation, d’intégration et de réussite pour les jeunes filles, nous proposons qu’un rapport soit remis au

Nous considérons que cet article est déjà satisfait et c’est pourquoi nous proposons de le supprimer. Il empiète sur les compétences du maire, qui a déjà l’autorité nécessaire pour encadrer ou interdire un rassemblement religieux si celui ci trouble l’ordre public, la tranquillité ou la sécurité Autrement dit, cette disposition transgresse les pouvoirs de police du maire et risque même de créer une confusion juridique. Elle ouvre la porte à des interprétations floues et à des contentieux inutiles. Elle ajoute une contrainte excessive qui pourrait conduire à des décisions profondément discriminatoires.

Il s’inscrit aussi en opposition avec l’esprit de la loi de 1905 et la jurisprudence du Conseil d’État, qui autorise la mise à disposition de locaux communaux au profit d’une association cultuelle, à condition qu’il ne soit pas transformé de façon exclusive et définitive, sans contrepartie financière, en édifice cultuel.

présenter l’amendement n° 12. Cet article interdit l’usage exclusif d’un équipement sportif à des fins cultuelles, mais cet objectif est déjà pleinement garanti par la jurisprudence. Le Conseil d’État, de manière constante, rappelle que, si une collectivité peut ponctuellement autoriser l’utilisation d’un équipement public pour l’exercice d’un culte, elle ne peut en aucun cas en accorder l’usage exclusif ou pérenne. Cet article, inutile juridiquement, est très révélateur de l’esprit de cette proposition de loi : il s’agit de détourner le principe de laïcité à des fins politiques et surtout discriminatoires. Quel était l’intérêt d’inscrire notamment comme salle de prière collective » dans cet article ? Nous demandons donc sa suppression. Nous demandons également la suppression de cet article. Le droit actuel est suffisant pour préserver la neutralité des locaux de tout contournement,

prévus dans la convention de mise à disposition location du bien pour faire respecter les engagements de l’association. La parole

parce que je suis partisan d’une application stricte de la loi de 1905. Ensuite, je signale à votre attention l’existence de la Fédération sportive et culturelle ; cette association sportive chrétienne, qui se revendique comme telle, s’emploie à développer la pastorale par le sport. Elle dispose d’aumôniers, nommés par la Conférence des évêques de France ; or je suppose que, s’il y a des aumôniers, c’est pour qu’ils aillent jusque dans les vestiaires.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain.

Il convient au contraire de faire monter en charge les outils existants, de mieux les faire connaître auprès des associations sportives et d’augmenter le nombre de contrôles. C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe RDPI propose de supprimer cet article 2 , qui est déjà satisfait par le droit existant.

lorsque celle ci est reconnue coupable de discrimination au sens de l’article 225 1 du code pénal. Vous proposez, monsieur le rapporteur, qu’une association sportive perde son agrément si certains de ses membres portent un signe religieux ou politique en compétition, alors même que cela ne relève ni d’une infraction pénale ni d’une atteinte au bon fonctionnement du sport. En revanche, une association condamnée pour discrimination raciale, sexiste ou homophobe pourra continuer à bénéficier de son agrément et de ses aides publiques. Cette incohérence est inacceptable ! Comment justifier que l’expression d’une croyance religieuse soit plus sévèrement réprimée que des actes de discrimination avérés ? Plutôt que de stigmatiser, nous devons mettre la lutte contre les discriminations au cœur des priorités du monde sportif.

du code du sport, le préfet « suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a

« respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine », ce qui est incompatible avec la commission d’infractions de discrimination, et à « s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public », ce qui est aussi incompatible avec la commission de toute infraction.

entre la neutralité du service public, qui concerne ses agents, et la liberté des usagers, qui peuvent exprimer leurs convictions tant que l’ordre public est respecté. Aujourd’hui, les autorités peuvent d’ailleurs déjà interdire une tenue pour des raisons d’hygiène d’hygiène ou de sécurité. De la sorte, cet article remet en cause l’équilibre de la loi de 1905, qui garantit à la fois la neutralité des institutions et la liberté de conscience des citoyens. Nous proposons donc d’adopter cet amendement de suppression de l’article 3, afin de préserver cet équilibre fondamental

Une telle mesure va à l’encontre du droit en vigueur, du principe de laïcité et de la libre administration des collectivités territoriales. Les principes de neutralité religieuse et de laïcité s’appliquent aux agents du service public et non à ses usagers. La parole

Lorsqu’il prend en compte pour l’organisation du service public les convictions religieuses de certains usagers, le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles

Il y en a un qui est oublié : le critère de respect des règles collectives. Je veux bien que, par la loi, on reprenne de façon presque intégrale la jurisprudence qui est en vigueur ; en revanche, ce qui est plus difficile à admettre, c’est que vous nous proposiez de placer cette

décision du 21 juin 2022, relative au règlement des piscines municipales de la ville de Grenoble. Le Conseil d’État a précisé à cette occasion que le gestionnaire d’un service public est tenu « de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l’égalité du traitement des usagers Autrement dit, la règle doit être la même pour tous. Il n’est pas possible de procéder à des adaptations pour un public particulier, notamment pour des raisons religieuses. Je rappelle que les dispositions de l’article premier de la Constitution interdisent en effet à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques

qui est tout à fait exceptionnelle. Les juristes nous expliquent que ce qui a motivé le Conseil d’État, ce n’est pas la loi de 1905, ce n’est pas la laïcité, c’est tout à fait autre chose : le respect des règles collectives et l’égalité de traitement des usagers du service

des événements qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre,… Exactement ! … des événements qui ont nécessité la sortie de l’ensemble des baigneurs, parce que la situation

d’ordre public ou d’hygiène. Depuis plusieurs années, certaines municipalités cherchent à interdire le port de tenues de bain couvrantes, notamment le burkini, sans que cela repose sur des impératifs d’hygiène ou des motifs d’ordre public. Le Conseil d’État lui même a rappelé en 2016 que ces interdictions portaient une atteinte grave aux libertés individuelles, en particulier à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté individuelle. Nous faisons face ici à une dérive inquiétante : des décisions administratives visent directement une partie de la population non pas pour des raisons de sécurité ou de santé publique, mais pour des considérations

Au moment où l’actualité ne cesse de mettre en exergue la dangerosité de l’islam radical sur notre territoire national, il est urgent de protéger dans les clubs sportifs nos plus jeunes concitoyens d’un quelconque

Par conséquent, il s’agit d’interdire à toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès des mineurs si elle est inscrite dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Quel est l’avis de la commission ?

qu’avec les services de plusieurs ministères engagés dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente. Seuls les destinataires habilités peuvent accéder aux données contenues dans ce fichier.

À l’article 4, nous envisageons de permettre la réalisation d’enquêtes administratives préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, comme c’est déjà le cas pour l’accès à certains emplois dans les domaines de la sécurité et de la souveraineté ou pour l’accès à des sites et événements particulièrement sensibles. L’enquête administrative doit permettre de détecter si la personne est habilitée à exercer son activité d’éducateur sportif auprès de jeunes enfants, mais, sans condamnation, il ne peut

Madame Lavarde,

l’épaule. Nous constatons aujourd’hui que, pour des raisons idéologiques, vous ne voulez pas voir que les choses ont évolué. Pour ma part, je remercie Michel Savin d’avoir proposé ce texte et je remercie le rapporteur

Elle va à l’encontre de notre Constitution, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle va à l’encontre du code du sport, qui garantit la liberté de pratiques sportives sans discrimination d’aucune sorte. Alors que le sport doit être un vecteur d’apprentissage de la citoyenneté, d’émancipation et de cohésion sociale, cette proposition de loi vient exclure de la pratique sportive des citoyens français. Elle risque en particulier d’éloigner les femmes portant le voile de la pratique sportive, alors que les femmes sont déjà plus éloignées du sport

portent le voile et subissent des discriminations tout au long de leur vie. La liste de ces discriminations est longue : agressions verbales, agressions physiques, discriminations lors de la recherche d’un logement, discriminations lors des contrôles de police, discriminations dans le monde du travail, que ce soit lors de la recherche d’un emploi ou tout au long de la carrière professionnelle. Par ailleurs, comment comptez vous appliquer cette loi dans les communes ou les départements majoritairement musulmans, par exemple Mayotte ? Voulez vous en faire des zones de non droit ? Les territoires où l’intégration et la cohésion sociale sont des réussites ne sont pas ceux où les communautés se sont montrées du doigt ou se sont tourné le dos. À La Réunion, je vous le redis, nous avons choisi le chemin du partage et de l’échange. Chez nous, la laïcité vit sans abîmer ni les identités ni les croyances. Nous refusons que la laïcité soit instrumentalisée par des lois aux relents de racisme et de sexisme. Ce n’est pas en participant à la stigmatisation d’une communauté que nous construirons une société apaisée et laïque ni que nous contribuerons à l’émancipation des citoyennes et des citoyens. Enfin, je tiens à vous dire que la voie assimilationniste n’est que le chemin de l’erreur.

Depuis plus de soixante ans, en effet, je fréquente les vestiaires en tant que pratiquant, dirigeant, père aussi.

Le scrutin est ouvert.